J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la mission d'information sur la réinsertion des mineurs enfermés a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. La parole

Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au et figurera dans l'analyse politique du scrutin. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour un nouveau pacte ferroviaire

Mais, sur le fond, en termes de coût global pour nos concitoyens, notamment compte tenu du recours à l'emprunt, la solution proposée n'est pas

Le scrutin est ouvert.

faire circuler des contre-vérités de nature à inquiéter les cheminots au moment où le Gouvernement envoie un message de confiance dans le transport ferroviaire, dans la SNCF et aux cheminots

maintenant. Ma réflexion est complémentaire. Il est essentiel de désendetter l'entreprise ferroviaire. Aucun système ferroviaire au monde n'est rentable seul, tant le monopole ouvert qu'il constitue nécessite

qu'il ne s'agit pas de remettre en cause aujourd'hui, tant les élus étaient nombreux dans l'ensemble des territoires à vouloir que ceux-ci soient desservis par le TGV. Force est de le constater, l'ensemble du réseau a souffert et s'est dégradé

à me convaincre de la pertinence et de l'intérêt du passage en société anonyme. Je considère que l'ensemble de la réforme que vous portez

dans la loi qu'on favorise la lutte contre le changement climatique en développant le fret ferroviaire. C'est bien, également, de mettre la réalité en conformité avec ses engagements.

Le scrutin est ouvert.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

provoquant une hausse des taux d'intérêt directeurs de 0,4 %. De plus, certains emprunts obligataires publics ne seraient plus possibles.

les gares ! Les explications, vous les avez ! Je pense que vous ne voulez pas les entendre.

Le scrutin est ouvert.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

qui sera responsable du domaine public ferroviaire national, et, d'autre part, l'opérateur public qui sera mis en concurrence avec d'autres opérateurs, le cas échéant. Il nous semble qu'il ne faut pas forcément traiter de manière symétrique SNCF Réseau et

l'idée de mieux garantir la présence des syndicats, des usagers et surtout des collectivités dans l'administration

Dans le prolongement de ce qui vient d'être dit par mon collègue Olivier Jacquin, je précise qu'il ne faut pas s'arrêter à l'exemple de la crèche, dont j'ai constaté qu'il faisait un peu réagir sur les travées de notre hémicycle. Ce qu'il faut retenir, c'est l'idée- elle me semble très

utile et même indispensable pour faire vivre l'idée que le service public, justement, c'est de la connexion entre les services publics, et pas chacun sur son rail

progressivement, au fur et à mesure que les transports se développent, devient la place du village, c'est-à-dire le lieu le plus fréquenté. C'est déjà le cas en Île-de-France ; c'est le cas aussi dans certaines

Dans les gares, des espaces destinés à des activités à but non lucratif sont réservés aux collectivités territoriales.

Madame la ministre, vous

les futurs embauchés ne seront plus au statut, et seront donc au régime de droit commun. Par ailleurs, vous le savez, une réflexion générale sur la pérennité de notre système de retraites a été confiée à Jean-Paul Delevoye. L'objectif est d'avoir un système qui maintienne la solidarité entre les générations et vise à plus de justice et d'équité,

de la réforme de la SNCF. Dès aujourd'hui, il y a un déficit démographique, qui, comme dans tous les secteurs, est compensé par la solidarité nationale. Notre réforme ne traite pas des retraites, ce sujet relevant de la réflexion globale conduite par Jean-Paul Delevoye.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos. J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement

Le scrutin est ouvert.

jusque-là, ça nous convient -« directement ou par l'intermédiaire de filiales ». Nous aimerions comprendre : comment peut-on réussir à défendre le service public

Nous estimons que la notion d'aménagement du territoire n'est pas claire, ou du moins qu'elle est trop vaste au regard du début de l'alinéa en question, qui précise que les missions sont exercées de façon « non discriminatoire En effet, promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique aussi peu précise permettrait de préparer les esprits à la fermeture de lignes qui pourraient être jugées insuffisamment rentables. Cela invite à mettre en balance la solidarité territoriale avec d'autres critères, comme celui de la rentabilité. C'est pourquoi nous préférons une formulation plus claire, pour que ces missions soient exercées dans une logique de solidarité nationale permettant de garantir le droit à la mobilité pour l'ensemble des territoires. Pour notre part, nous portons une vision tout autre de l'aménagement du territoire, fondée sur la solidarité et l'égalité de traitement pour un développement humain soutenable. soutenable. La SNCF ne remplit pas n'importe quelle mission : elle concourt d'une manière fondamentale à l'organisation cohérente de notre système de transports, avec l'objectif de répondre aux besoins en matière de transports et d'efficacité économique, sociale et environnementale, au service d'un aménagement du territoire équilibré, facteur de réduction des inégalités territoriales. En outre, le rôle du service public est de garantir le droit aux transports pour tous,

Déjà à l'époque, et sans surprise, nous avions voté contre cette disposition qui ouvrait une brèche dans l'unicité du réseau et la voie à son démantèlement. Nous sentions poindre, alors, l'idée du Gouvernement de se défausser des petites lignes, notamment sur les régions.

Le rapport Spinetta, en promettant l'abandon de 9 000 kilomètres de ligne, précipite ce scénario, puisque le maintien de ces lignes est renvoyé aux futurs contrats de plan. Nous pouvons vous croire quand vous parlez d'un effort particulier en faveur de ces contrats de plan, mais nous avons un sérieux doute. Et il ne s'agit

certaines missions relatives aux lignes à faible trafic. Cette faculté est pourtant intéressante, puisqu'elle permet, par exemple, à SNCF Réseau de confier à d'autres entreprises le soin d'assurer l'entretien ou la maintenance de petites lignes lorsque ses propres équipes sont mobilisées sur d'autres travaux. Le code des transports encadre cette faculté, puisqu'il précise que cette délégation ne peut concerner les missions de répartition des capacités et de tarification de l'infrastructure. En clair, l'adoption de cet amendement

Je partage l'avis de la commission. Le groupe du RDSE pourra vous réponde sur les intentions du Gouvernement dans la réforme de 2014. Effectivement, cet alinéa que vous voulez supprimer permet d'accélérer la rénovation du réseau ferré national. C'est un levier utilisé, par exemple, par la région Grand-Est pour redynamiser le fret ferroviaire. On ne peut pas tout à la fois vouloir défendre le fret ferroviaire et priver nos entreprises de la capacité de moderniser les réseaux. Avis défavorable.

Nous discutons depuis hier, et pour quelques jours encore, de la loi ferroviaire, puis appréhenderons à l'automne, me semble-t-il, la question plus large des mobilités.

plus largement des mobilités. Or le fait que la loi ferroviaire nous soit présentée aujourd'hui nous empêche d'appréhender un certain nombre d'autres aspects.

PPP. Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour SNCF Réseau de recourir à des contrats de concession ou de partenariat pour l'exercice de certaines missions. Personnellement, je ne suis pas un « fan » des PPP, mais je pense qu'il faut par moments laisser une certaine souplesse.

est regrettable d'abandonner l'ensemble de ces espaces à la consommation. La République française privilégie systématiquement le commun par rapport au particulier. Elle est un projet politique conscient et performatif de résistance à l'empiètement de la sphère privée sur la sphère publique, pour le bien de nos concitoyens. Seul l'État, normalement, a ce souci-là. La

Luxembourg, filiale qui permet à la SNCF d'alléger le montant de son impôt en France. Elle a été créée en octobre 2012. Elle est dotée de 11 millions d'euros dans le premier rapport financier qui a suivi sa création. Savez-vous combien elle a de salariés ? Un seul salarié entre dans la composition de cette entreprise, qui n'a d'ailleurs qu'une boîte postale dans un immeuble du duché du Luxembourg. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas le montant financier total confié à cette filiale, mais nous connaissons son fonctionnement

qui ne sont pas très respectés depuis deux mois, et les Français, qui financent l'ensemble du système ferroviaire. Ce sont ces trois groupes qui doivent avoir la parole. Je ferai quatre réflexions.

constituent une avancée. La reconnaissance des gares comme un élément du système ferroviaire qui mérite une concertation avec les acteurs figure dans cet article. Je m'en réjouis.

Madame la ministre, nous en avons parlé plusieurs fois, c'est un véritable sujet. Nous avons besoin de vous entendre nous confirmer, même si vous l'avez déjà dit plusieurs fois, que les contrats de plan continueront à porter ces investissements et qu'ils seront honorés et réalisés. En effet, le problème vient de la non-réalisation dans le passé des contrats de plan.

quinze heures sous le titre : « La patronne de la RATP défend le statut public de l'entreprise de transport ». Je cite un extrait : « Lors de la présentation de ses résultats 2017, vendredi 23 mars, la nouvelle [présidente de la RATP] a clamé son attachement au statut public de son entreprise et à celui de ses agents. » La présidente de la RATP l'assure : « Être un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), directement sous la tutelle souvent embrouillée de l'État, ne handicape en rien la RATP. » Ces affirmations ont été reprises samedi, sur France Inter, où la présidente de la RATP a bien précisé que ce statut pouvait même convenir pour affronter la concurrence. Voilà quelques éléments

d'une infrastructure qui irrigue l'ensemble du territoire et qui réponde aux différents usages du ferroviaire, que ce soit pour les marchandises

Il faut savoir raison garder dans les arguments, sinon on tombe dans les excès. La plupart de nos gares dans notre pays ne relèvent pas de projets pharaoniques. Il faut simplement redonner de la vie et de l'utilité à l'ensemble des gares pour que nous puissions encore les fréquenter demain.

dans l'intérêt des voyageurs, de la SNCF et des cheminots.

Ce texte apporte un certain nombre de garanties. Il est clair qu'il répond au souhait de la majorité de la représentation nationale : garanties financières dans le domaine de la dette, dont la SNCF était en grande partie non responsable, garanties en matière de développement durable, garanties sur la desserte des territoires, garanties pour les usagers.

notamment au travers de l'article 1 A, n'offre aucune garantie. Ce ne sont, depuis le début, que des paroles. Quand on les met en doute, on est accusé de caricaturer la politique du Gouvernement. Je veux le redire ici

desserte de l'ensemble du territoire par un service ferroviaire de grande qualité. Madame la ministre, depuis le début, vous ne répondez à aucun de ces sujets. Vous affirmez simplement

Le scrutin est ouvert.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

La séance est suspendue.